Nous reprenons l'examen de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à agir contre les violences au sein de la famille. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre I, à l'article 2. La parole est à Mme Laurence Cohen,

La lourdeur administrative est en partie responsable de cette faible délivrance. L'une des principales dispositions prévues dans l'article 2, à savoir la réduction des délais de délivrance à six jours maximum à compter du jour de la fixation de l'audience, permet de redonner son utilité première à l'ordonnance étant, pour nous- c'est l'objet de l'amendement n° 29, que je défendrai dans quelques instants -, il serait préférable de fixer le délai à compter de la requête de la victime. Bien entendu, cela suppose que la justice ait les moyens d'accomplir ses missions.

électronique. La demanderesse aurait une sorte de boîtier. Ainsi, en fonction d'une distance imposée par le juge, il n'y aurait pas de possibilité de rapprochement physique pendant une durée fixée par lui.

très ingénieuse, qui consiste à doter le juge des affaires familiales d'une palette de prérogatives pour répondre à une situation de danger pour une personne victime de violences au sein de son couple. Selon les données disponibles, dans un cas sur deux, la demande d'ordonnance serait rejetée, en partie du fait de la difficulté d'établir l'existence de « raisons sérieuses » de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger. et le danger. Compte tenu des moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales, le législateur s'est montré très précautionneux dans sa rédaction, ce qui rend l'ordonnance plus difficilement applicable. applicable. En vue de mieux protéger les éventuelles victimes, nous proposons que l'ordonnance de protection puisse être plus facilement délivrée en supprimant la référence aux « raisons sérieuses », afin de laisser une plus large interprétation au juge. En contrepartie de cet élargissement, nous serions favorables à ne pas multiplier les moyens coercitifs conférés au juge des affaires familiales par le biais de l'ordonnance de protection et à ne pas étendre le recours du bracelet anti-rapprochement à ce cas de figure précis.

En outre, du fait de la nature hybride de l'ordonnance de protection, la procédure qu'il est proposé d'instaurer n'offre pas à la victime la garantie formelle de l'éloignement. Admettons par exemple que l'auteur présumé de violences refuse le port du bracelet anti-rapprochement et soit condamné à la peine prévue par ailleurs. A-t-on la certitude que la sanction sera automatiquement prononcée et exécutée ? L'individu sera-t-il effectivement incarcéré ? Pour combien de temps ? Et qu'adviendra-t-il, le cas échéant, à sa sortie de prison ? Nous vous proposons donc un nouvel équilibre de l'ordonnance de protection, fondé sur un élargissement de son application à moyens constants pour le juge.

heures, afin de tenir compte de l'urgence qui s'attache à la protection du conjoint victime et, le cas échéant, des enfants du couple. Bien évidemment, ayant entendu ce qui s'est dit lors de la discussion générale, je sens bien que le délai de trois jours est absolument impossible à tenir. Mais, vous le comprendrez, il s'agit d'un amendement d'appel.

répondant mieux à la nécessité d'une mise en sécurité durable et efficace d'une femme victime de violences. Nous nous inscrivons dans une démarche de principe de précaution. C'est la raison pour laquelle nous proposons de réduire les délais à six jours maximum, mais à compter de la requête de la victime. À notre avis, cela va

et que la mesure soit prononcée en dehors de toute poursuite pénale. Le juge aux affaires familiales ne saurait en effet ordonner une telle mesure dans le cadre d'une procédure civile où il n'est question que de « faits de violence allégués ». Il s'agit d'une prescription attentatoire aux libertés individuelles. Elle doit nécessairement rester de la compétence du juge pénal, après examen et débat contradictoire sur les charges pesant sur l'intéressé.

qu'il faut recueillir l'accord du défendeur, afin de ne pas se trouver face à un problème constitutionnel d'atteinte à la liberté d'aller et venir, puisque nous sommes en phase pré-sentencielle.

n'a pas la compétence d'instaurer des mesures restrictives de liberté de cet ordre. Nous voyons donc bien qu'il y a là une difficulté conceptuelle. Il faudrait se rapprocher de la compétence du juge pénal.

une proposition : lorsque le juge aux affaires familiales envisage de demander un bracelet anti-rapprochement, il saisit le ministère public, qui peut demander au juge des libertés et de la détention, dont c'est le métier,

pas les modalités précises. D'un point de vue purement juridique, le dispositif pose également question. Les placements sous surveillance électronique relèvent aujourd'hui de la compétence dévolue au juge pénal, dans le cadre de la procédure pénale. Avec cet article, le juge aux affaires familiales pourra, dès la délivrance de l'ordonnance de protection, prévoir un placement sous surveillance électronique mobile de l'auteur présumé de violences conjugales, alors que l'affaire n'aura pas encore été jugée au fond, mais seulement Nous considérons pour notre part qu'une telle mesure, aussi attentatoire aux libertés individuelles, doit être prononcée par le juge pénal, après examen des charges pesant sur l'intéressé C'est également ce que relève le Conseil national des barreaux, pour qui le JAF « ne saurait ordonner une telle mesure alors que le dispositif est prévu dans le cadre d'une procédure civile où il n'est question

alors le juge des libertés et de la détention, lequel pourra ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port, par chacune d'elle, d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement. Il s'agit d'être rigoureux dans l'application de telles sanctions, surtout lorsqu'elles sont prononcées prononcées à titre pré-sentenciel. Les grands principes de notre droit doivent demeurer, quelle que soit la gravité du sujet traité.

En premier lieu, il vise à assouplir les conditions de délivrance de l'ordonnance de protection, en supprimant les « raisons sérieuses » sur lesquelles le juge doit aujourd'hui se fonder pour estimer la vraisemblance des faits de violences allégués. Cela ne me semble pas du tout opportun, car l'ordonnance de protection n'est qu'une mesure provisoire, adoptée au terme d'une instruction très réduite. La décision du juge civil repose sur la plausibilité des violences et du danger. Dès lors, il est primordial d'exiger qu'il se prononce sur la base d'éléments sérieux, sauf à risquer de porter gravement atteinte à la présomption d'innocence. Nous sommes donc très opposés à la suppression du critère des « raisons sérieuses

Nous pensons toutefois que l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le prononcé de la mesure ne constituerait qu'une garantie d'affichage, le cadre juridique n'étant toujours pas,, celui d'une procédure pénale. Dès lors, même si le JLD pouvait se passer du consentement du défendeur pour ordonner le port du bracelet, la « pose » de celui-ci ne pourrait être effectuée sans son consentement,

, présenté par Laure Darcos, tend à réduire à trois jours le délai dans lequel l'ordonnance de protection est délivrée. Calqué sur le modèle espagnol, le délai de 72 heures semble déjà très court pour permettre aux juridictions de se prononcer en respectant les exigences du contradictoire. demeurant, la comparaison qui est faite régulièrement avec le modèle espagnol n'est pas complètement pertinente, l'Espagne ayant créé des juridictions spécialisées en matière de violences conjugales- nous y reviendrons peut-être, madame la garde des sceaux -composées de juges disposant de prérogatives en matière pénale et civile. Toute tentative de transposition se heurte donc à des difficultés un peu lourdes, auxquelles la proposition de loi a tenté de remédier en imposant un délai de six jours, déjà bien plus court que le délai moyen actuel de

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale permet de conserver ce délai de six jours, tout en laissant au magistrat une plus grande souplesse

pénal. La définition actuelle des violences inclut donc bien les violences psychologiques mentionnées à l'article 222-14-3 du code pénal. À cet égard, le guide de la Chancellerie mentionne explicitement les violences psychologiques, avec les violences sexuelles ou physiques, comme susceptibles de relever de l'ordonnance

par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien entendu, le défendeur doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense, ce qui me semble assez difficilement compatible

peut être caractérisée même lorsque les parties ne vivent pas sous le même toit. J'émettrai un avis de sagesse sur cet amendement, dont je comprends évidemment le sens.

le bracelet anti-rapprochement, qui peut être prononcé à différents stades de la procédure civile- en pré-sentenciel, pendant le contrôle judiciaire ou en post-sentenciel -, ne constitue ou en post-sentenciel -, ne constitue pas une peine au sens pénal du terme, qui serait prononcée à l'encontre de l'auteur des faits. Il s'agit en réalité d'une mesure de protection envers une victime en danger.

Bien sûr, les raisons de cette faible réussite sont multiples et peuvent découler aussi du découragement des parties demanderesses. Toutefois, la difficulté de prouver l'existence de violences vraisemblables paraît excessivement dissuasive. En parallèle, nous savons qu'il existe un certain nombre de dysfonctionnements dans les systèmes d'alerte et que les signaux faibles des violences familiales ne sont pas utilisés comme il le faudrait. Ainsi, les personnels des hôpitaux et de l'éducation nationale qui en constatent les stigmates sur les corps des enfants ou des femmes, en particulier celles qui sont suivies pendant leur grossesse, moment de vulnérabilité vulnérabilité toute particulière, éprouvent parfois des difficultés à agir au secours de ces personnes. Nous savons que des propositions sont à l'étude, notamment la possibilité de déposer plainte à l'hôpital- cette possibilité pourrait être étendue aux infirmeries scolaires. Là encore se pose une question budgétaire importante. Nous proposons donc une solution alternative qui permettrait de mettre en contact le JAF, chargé de l'ordonnance de protection, et ces témoins de violences ou de leurs effets, afin qu'ils puissent utilement contribuer à la sécurisation des victimes. Quel est l'avis de la commission ?

travaillant dans une unité hospitalière spécialisée, par un chef d'établissement scolaire ou par une infirmière scolaire. Il est vrai que les professionnels de santé et les personnels de l'éducation nationale sont bien placés pour repérer les situations de violences intrafamiliales, dont peuvent être victimes les femmes et les enfants. Un signalement effectué par l'un de ces professionnels est un élément d'appréciation important, qui mérite d'être porté à la connaissance du juge. Il me semble cependant que l'on ne peut pas donner à ces signalements les effets juridiques envisagés par l'amendement. En effet, tous les éléments du dossier doivent être débattus c'est un principe fondamental qui découle du droit à un procès équitable. On ne peut donc pas considérer que les violences ou le danger sont établis dès le stade du signalement. Un professionnel peut procéder à un signalement, parce qu'il a un doute

Le scrutin est ouvert.

que, à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur plusieurs mesures. De fait, cette rédaction rend facultative la décision de statuer sur telle ou telle mesure de protection permise par l'ordonnance. Cet amendement a pour objet de renforcer l'efficacité de l'ordonnance de protection. proposons que le juge statue effectivement sur chacune des mesures ouvertes dans ce cadre. Cela peut être nécessaire notamment pour les mesures relatives aux enfants à l'autorité parentale et pour celles permettant à la victime de dissimuler son identité, mais aussi pour ce qui concerne le logement ou l'interdiction pour le défendeur de recevoir ou de rencontrer des personnes, autant de mesures qui peuvent parfois ne pas être étudiées par le juge, alors qu'elles pourraient s'avérer utiles, pour ne pas dire

pose des difficultés, puisque, en principe, le juge civil ne peut statuer que sur des demandes qui ont été formulées et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire. Le texte adopté à l'Assemblée nationale et conservé par notre commission des lois a permis d'aboutir à un point d'équilibre entre ce que la procédure permet et le souhait de voir le juge se prononcer davantage sur le panel des mesures de l'ordonnance de protection. Lors de l'audience, le juge qui dirige les débats demandera aux parties si elles ont des observations sur tel ou tel point afin de pouvoir en être saisi et, le cas échéant, ordonner une des mesures,

le juge « se prononce sur chacune des mesures suivantes » porterait davantage atteinte au contradictoire que la rédaction actuelle, selon laquelle le juge « est compétent ». Je ne crois pas que ce soit le bon argument

a adopté plusieurs amendements tendant à imposer au juge des obligations supplémentaires de motivation. Cela ne me semble pas pertinent au regard de l'obligation de motivation générale qui pèse déjà sur les juges pour tout jugement. par cet amendement, de revenir sur l'obligation de motivation spéciale en cas de refus de prononcer l'interdiction de port d'arme, lorsqu'une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les enfants est prononcée.

par définition, de motiver sa décision. L'obligation de motivation spéciale m'apparaît donc sans objet. J'ajoute que, sur ce sujet précis des armes, ce qui compte, c'est l'effectivité de l'interdiction d'acquérir ou de porter une arme. C'est pour cette raison que je vous proposerai tout à l'heure un amendement permettant d'inscrire cette interdiction dans un fichier.

je ne vois donc pas de difficulté particulière. Le principe de la motivation spéciale existe en droit civil et est fréquent en droit pénal. Je ne crois donc pas que cela affaiblisse le principe général de motivation. La commission émet donc un avis défavorable

laisser à son conjoint violent. Nombre de victimes quittent leur domicile ou acceptent devant le juge aux affaires familiales de le faire pour mettre fin à une situation qui dure depuis trop longtemps et, ainsi, pour se mettre à l'abri. Dans l'urgence, il s'agit bien de cela

; il est très déstabilisant d'être dans une itinérance forcée, le temps que le délai soit accordé au mari de quitter le domicile ou que l'affaire soit réglée.

Outre le fait qu'il ne concernerait que les époux et non les partenaires de PACS ou les concubins, ce qui pose déjà un problème d'égalité, cet amendement ne me semble pas opérationnel. L'attribution de la jouissance du logement à la victime de violences est le principe, si la victime en fait la demande. En outre, l'article 515-12 du code civil répond déjà à votre demande. Il permet en effet que le juge prenne de nouvelles mesures, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une des parties. La victime pourra, dans ce cadre, formuler la demande d'attribution du logement qu'elle n'aurait pas formulée initialement. Elle a le droit de changer d'avis ! La commission demande donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait par le droit en vigueur.

le bailleur ne pouvant rompre celui-ci qu'avec l'accord exprès de la victime qui occupe le logement. Ainsi, l'ordonnance de protection produirait des effets opposables au propriétaire bailleur du logement occupé par la victime

ou conjugal ». Or les époux sont automatiquement cotitulaires du bail : dans cette hypothèse, aucune résiliation unilatérale du bail n'est possible. Les partenaires d'un PACS peuvent également être cotitulaires du bail, s'ils l'ont demandé, mais cela n'est pas automatique. La disposition que vous proposez ne peut être applicable envers le bailleur : celui-ci n'a pas connaissance des décisions judiciaires et, surtout, il n'a aucune relation contractuelle avec la personne qui n'est pas titulaire du bail. En tout état de cause, une personne victime de violences à laquelle le JAF attribuerait la jouissance du logement ne pourrait pas être expulsée du logement, cette mesure ne pouvant être prononcée que par un juge. La victime bénéficiaire d'une ordonnance de protection ne serait pas considérée sans droit ni titre, et il n'est pas imaginable qu'un

des associations que nous avons entendus en amont de l'examen de ce texte nous ont décrit de nombreuses situations où l'auteur des violences organise son insolvabilité pour faire perdurer une forme d'emprise sur sa victime et la maintenir dans une situation difficile. Afin d'éviter ce cas de figure, il serait souhaitable que le JAF puisse se prononcer sur la possible désolidarisation des dettes liées à un crédit immobilier, sous réserve, bien entendu, de l'acceptation de la banque. Cette disposition rendrait trois services majeurs aux victimes de violences conjugales. Tout d'abord, celles-ci seraient informées de cette faculté, qu'elles ignorent bien trop souvent. Par ailleurs, elles pourraient justifier et appuyer leur demande auprès de leur établissement bancaire. Enfin, les situations d'organisation d'insolvabilité par un auteur de violences conjugales pourraient être prévenues.

pas très bien mesurés. S'il s'agit de prévoir que la victime ne rembourse pas sa part de l'emprunt pendant la durée de l'ordonnance de protection, cela ne signifie pas pour autant qu'elle serait libérée de la charge de la dette. Qu'en serait-il ensuite de la propriété du logement ? En revanche, ce qui est certain, et cela répond peut-être mieux à votre attente, c'est le droit en vigueur, confirmé par la proposition de loi. En effet, lorsque le JAF attribue la jouissance du logement à la victime, il peut aussi mettre à la charge du conjoint violent les frais afférents à ce logement.

du fait de leur rôle de témoins, soit directement, étant eux-mêmes victimes de coups. En outre, tous les rapports d'expertise établissent un lien clair entre la violence subie au moment du développement d'un enfant et le futur comportement de ce dernier en tant qu'adulte. Sans que la causalité soit absolue, il est courant que les enfants élevés dans des contextes familiaux violents deviennent à leur tour des adultes violents ou violentés. Pour tous, y compris ceux qui parviennent à s'extirper de tels climats, l'accès à la parentalité est difficile, par peur de reproduire ces schémas, à juste En mai 2018, l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale de la justice et l'Inspection générale de l'administration ont produit un rapport faisant suite à la mission sur les morts violentes d'enfants au sein des familles. au sein des familles. La recommandation n° 10 de ce rapport vise le renforcement du suivi par le juge des rencontres intermédiées entre parents et enfants, quand le climat familial est violent, en prévoyant une obligation de compte rendu. Tel est l'objet de cet amendement, appliqué au seul cadre de l'ordonnance de protection. Quel

au fond sur les modalités. La décision de ne pas prononcer la suspension devrait être spécialement motivée. Le juge peut déjà apprécier les modalités d'exercice de l'autorité parentale dans le cadre de l'ordonnance de protection et, par exemple, prononcer le retrait total ou partiel de ladite autorité, sur la base de l'article 378-1 du code civil. L'ordonnance de protection est déjà un jugement au fond, même si les mesures sont provisoires. La suspension de l'autorité parentale n'est, en outre, en l'état,

de permettre au JAF de solliciter un compte rendu du détail des rencontres entre parents et enfants, lorsqu'il ordonne un droit de visite dans un espace de rencontre ou avec l'assistance d'un tiers de confiance. L'intention est louable, mais cette disposition ne paraît pas très opérationnelle

civil. J'ajoute que ce sujet est traité dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. Mon collègue Adrien Taquet réfléchit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et des évolutions seront peut-être proposées à l'issue du Grenelle.

le même. Ainsi, en fonction de ce qui est signalé, le juge peut modifier sa décision initiale sur demande des parties, ou même d'office, ce qui est une exception aux règles ordinaires. L'esprit de votre amendement est respecté, et je serais heureuse que vous le retiriez. La

le 3 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé qu'allait être envisagée la possibilité de la suspension de l'autorité parentale en cas de violences conjugales.

indispensable dans le cadre de mesures provisoires, sachant que le juge sera amené, très peu de temps après, peut-être à l'issue d'une médiation, à trouver une solution pour que les relations entre les enfants et leur père puissent reprendre dans un contexte clair et rassurant pour tout le monde.

même tout à fait essentiel ! En revanche, lorsque vous évoquez les questions liées à la suspension de l'autorité parentale, vous posez là un vrai sujet. J'ai dit simplement

La question de l'autorité parentale est traitée très sérieusement dans ces groupes de travail. Je le rappelle, l'article que nous examinons précise expressément que le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut donc, dans ce cadre, attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un

Le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Quand il délivre son ordonnance de protection, le JAF peut donc déjà retirer l'autorité parentale. Ne pensons pas qu'il ne peut rien faire ! Cette possibilité est déjà prévue dans le code.

Il s'agit de retirer à l'un des parents l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale. Il n'est donc pas possible de le faire si le juge ne retire pas l'autorité parentale au défendeur à une ordonnance de protection. Eh bien, voilà, Les deux sont liés : si le juge confie l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des deux parents, alors, il est possible de le priver de certaines informations relatives à la vie quotidienne et à l'éducation de l'enfant. On a compris ! Je sais bien que vous avez compris, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je me permets donc de redonner les explications Alors, tout le monde a compris qu'on essaye de faire au mieux ! Cela étant dit, la nouvelle interdiction de paraître que prévoit la proposition de loi permettra, le cas échéant, d'interdire au défendeur de se rendre dans le périmètre de l'école des enfants si le juge l'estime nécessaire. C'est donc un avis défavorable.

rester sur vos rails, rien que sur vos rails. L'initiative doit venir de votre part, à un moment qui sera utile pour votre communication, autour du 25 novembre, une date emblématique. Je ne partage pas cette façon de faire parce que les victimes vont rester dans le dénuement

parce que l'autorité parentale se décide dans le cabinet du juge. Elle peut être retirée, accordée, exclusive, partagée,

il est impossible de traiter les violences faites aux femmes en se limitant à une ou deux mesures. Moi non plus, je ne comprends absolument pas la volonté de s'opposer systématiquement à ces amendements qui sont le fruit du terrain. La délégation aux droits des femmes

515-11 du code civil. Dans son dernier alinéa, il était prévu que lorsque, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales était amené à considérer que des enfants étaient en danger, il devait prévenir le procureur de la République. Nous proposons de supprimer cette indication « en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants », considérant que le juge doit d'office informer le procureur de la République de l'ordonnance de protection qu'il prend. Cela paraît d'autant plus indispensable que le même texte prévoit que le dépôt de plainte n'est plus nécessaire au dépôt de la demande d'ordonnance de protection. la démarche peut être faite devant le juge aux affaires familiales sans que le procureur de la République soit informé d'un délit qui est commis à l'égard d'une femme.

dans tous les cas, l'ordonnance de protection est communiquée au procureur de la République, à charge pour lui de faire une enquête et de suivre. Si nous voulons protéger les victimes, cette démarche est indispensable. Quel est l'avis de la commission ? de la commission ? Le présent amendement tend à informer le procureur de la République de toutes les ordonnances de protection qui sont délivrées. Il est déjà satisfait par le droit positif. à tous les stades de l'instance civile. Il reçoit toutes les demandes d'ordonnance de protection et est partie jointe à l'audience dans la plupart des cas. Enfin, il est informé des suites données à toutes les demandes d'ordonnance de protection, puisque la décision prise par le juge aux affaires familiales lui est notifiée pour information par remise avec émargement ou envoi contre récépissé. Il doit procéder à l'inscription au fichier des personnes recherchées, des personnes faisant l'objet d'une interdiction de contact ou de détention et de port d'armes et, bientôt, de celles qui feront l'objet d'une interdiction de paraître. Le juge aux affaires familiales effectue en outre auprès de lui un signalement spécifique sans délai de toute ordonnance de protection délivrée en raison de violences susceptibles de mettre en danger

tout de même ... -pour tendre vers un seul objectif : trouver le meilleur dispositif pour lutter contre les violences conjugales. Ce texte est arrivé au Sénat dans des conditions invraisemblables.

vous. M. Buffet n'aura plus besoin de demander des scrutins publics ; vous pourrez voter ou non les amendements qui vous conviennent et nous n'aurons plus besoin de développer les arguments que nous tentons de vous faire entendre. Vous assumerez ainsi la responsabilité de ce travail parlementaire bâclé qui avait pourtant si bien commencé à l'Assemblée

au regard de la situation de la victime. Dès lors que cette dernière introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal ou le juge civil, l'ordonnance de protection, une fois obtenue, ne permet pas de la protéger jusqu'à l'aboutissement des procédures.

de violence est toujours présente. Actuellement, la deuxième phrase de l'article 515-12 du code civil ne vise la possibilité de prolongation de l'ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales que si la victime introduit une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l'exercice de l'autorité parentale. Or ces hypothèses ne couvrent pas les situations des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré. L'objectif de cette modification demandée par de nombreux acteurs est donc de renverser la logique et d'accroître la protection accordée aux bénéficiaires d'une ordonnance, afin de simplifier leur parcours, souvent fait de différentes procédures.

à six mois ce délai. Les mesures de l'ordonnance de protection peuvent également être prolongées au-delà de cette période si une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée ou si le juge a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale pour la durée de la procédure. Nous considérons qu'il s'agit d'un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l'atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent entraîner, sur la base de faits vraisemblables, par exemple, la nouvelle interdiction de paraître introduite par la proposition de loi. de loi. Si cet amendement était adopté, les mesures d'une ordonnance de protection pourraient ainsi être prononcées pour une durée indéterminée, ce qui me semble peu acceptable. L'ordonnance de protection est un outil d'urgence

Dans ce cas, il est proposé de rendre le juge compétent pour prendre les mesures mentionnées au nouveau 1° , à savoir l'interdiction pour l'auteur des faits de se rendre dans certains des lieux fréquentés habituellement par la victime. Quel est l'avis de la commission Cet amendement vise à étendre l'interdiction de paraître aux défendeurs à une ordonnance de protection en cas de mariage forcé. Le juge aux affaires familiales peut en effet délivrer une ordonnance de protection aux personnes majeures menacées

parole est à Mme Laure Darcos. Je souscris au principe du retrait du droit d'hébergement du conjoint violent, pour une durée déterminée, qui ne conserve qu'un droit de visite encadré, sauf à ce que le juge motive expressément son refus de prononcer cette mesure au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est toutefois proposé que ce droit de visite encadré s'exerce, non pas dans un simple espace de rencontre, mais dans un lieu protégé, en présence d'un tiers permettant d'assurer la continuité des relations sans mise en danger de l'enfant.

Mme Françoise Cartron. L'article 2 prévoit que le juge peut enjoindre les parents à consentir à une procédure de médiation familiale, sauf si des violences sont alléguées par l'un d'entre eux sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cet article est bienvenu dans la mesure où le rapport d'emprise asymétrique entre l'agresseur et sa victime peut conduire cette dernière à consentir, contre son gré, à la médiation. Toutefois, le principe d'interdiction de la médiation en cas de violence alléguée nous semble peu conforme aux garanties de la présomption d'innocence. Nous estimons en effet que la mesure de médiation relative à l'exercice de l'autorité parentale que le juge est susceptible de proposer peut être exclue lorsque celui-ci estime vraisemblable la commission de faits de violence. outre, la proposition de rencontrer un médiateur familial pourrait aussi être exclue lorsque les faits de violence commis par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant sont avérés et non seulement allégués. allégués. Quelle que soit l'option retenue, nous devons pouvoir faire l'économie d'une telle précaution législative en capitalisant, comme il se doit, sur l'appréciation discrétionnaire du juge. Les magistrats savent mieux que personne qu'une procédure de médiation entachée de violence est nulle et non avenue.

En réalité, ce changement n'aurait pas vraiment de conséquences, dans la mesure où cette interdiction n'est pas subordonnée à une condamnation ou à un dépôt de plainte. Seul le juge apprécie la situation. La Chancellerie, dans sa circulaire d'application de ces dispositions, indique déjà aux juges qu'ils devront apprécier s'il existe des faits de violence allégués. Pour ces raisons, la commission est défavorable

que toute personne ayant fait l'objet d'une ordonnance de protection était interdite de port et de détention d'armes, même si le juge aux affaires familiales ne l'avait pas ordonné, car cela était excessif. Cet amendement vise non pas à rétablir les dispositions supprimées, mais à les remplacer par d'autres prévoyant

Ce fichier peut être consulté par différentes administrations comme la police, la gendarmerie, les douanes, mais également par la Fédération nationale des chasseurs, les fédérations de tir sportif et les armuriers. Cet amendement permet donc de rendre effectives les interdictions qui ont été prononcées par le juge aux affaires familiales. Je précise, pour répondre à des interrogations qui ont été formulées ce matin en commission par Mme la rapporteur et qui expliquent - j'anticipe peut-être un peu ce que va dire Mme la rapporteur -l'avis de sagesse de la commission,

par le JAF, il vise à insérer dans ce même code un nouvel article L. 312-3-2 rappelant l'existence de ces interdictions. Quant à l'article L. 312-16, il renvoie lui-même à ce nouvel article.

constitue bien un délit de violation de cette ordonnance prévue par l'article 227-4-2 du code pénal. Cette pénalisation est en effet absolument indispensable pour assurer l'efficacité de la réforme. les forces de l'ordre ne disposeraient d'aucune base légale pour intervenir si l'auteur des violences se rapproche de la victime à moins d'une certaine distance fixée par le JAF, tant qu'il ne sera pas en contact avec cette dernière. Elles ne pourront que rester passives lorsque le dispositif générera des alertes. Ces dernières auraient ainsi pour seule conséquence d'informer la victime que l'auteur des violences se rapproche d'elle et qu'elle doit se mettre en sécurité, ce qui n'est pas, vous en conviendrez, l'objectif recherché. L'existence d'une infraction est donc juridiquement nécessaire pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir dans le cadre de l'enquête de flagrance, afin d'interpeller l'auteur et de le placer en garde à vue, avant que le procureur ne se prononce sur d'éventuelles poursuites. Le but n'est évidemment pas d'emprisonner la personne, mais de l'empêcher de se rapprocher de la victime. La situation justifie par conséquent de préciser la rédaction des dispositions de l'article 227-4-2 du code pénal, ce qui fait l'objet du présent amendement. Je précise que ce dernier a été rectifié,

dans son ordonnance de protection. J'espère que cette rectification conduira la rapporteur à émettre un avis favorable

le dispositif du bracelet électronique anti-rapprochement dans le cadre d'une ordonnance de protection qui s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2022, et que le Parlement devra à cette date pérenniser ou non. Pour autant, il paraît nécessaire d'en pénaliser la violation. En effet, En effet, même si le dispositif est adopté de façon temporaire par le Parlement, il doit bien évidemment être efficace. Or, si vous ne prévoyez pas de pénalisation, tel ne sera pas le cas. Je le répète, si on ne crée pas un délit de non-respect de la distance, les forces de l'ordre ne pourront pas intervenir lorsque l'auteur de la violence se rapprochera de la victime, tant qu'il ne sera pas en contact avec elle. Il me semble qu'il ne sert à rien d'instituer un dispositif anti-rapprochement si celui-ci ne permet pas d'empêcher effectivement ce rapprochement. S'il permet uniquement de prévenir la victime que l'auteur des violences se rapproche, que penseront les victimes du dispositif adopté par le Parlement ? Le but, je le répète, est de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir et d'intercepter la personne

visant à protéger les descendants. Cet amendement vise à modifier le code civil pour prévoir, à l'article 379, la dispense de l'obligation d'aliment pour l'enfant en cas de retrait total de l'autorité parentale ; rendre irrecevable la demande de restitution de l'autorité parentale prévue à l'article 381 du code précité, quand le parent qui en fait la demande a été condamné pour le meurtre ou l'assassinat de l'autre parent ; ; exclure l'obligation d'aliment des enfants à l'égard de leurs ascendants, définie par l'article 205 du même code, en cas de condamnation pour le meurtre ou l'assassinat de l'autre parent ;

en tout ou partie lorsque celui-ci a gravement manqué à ses obligations envers lui, ce qui semble évident s'il a tué sa mère. Mais cela suppose une action en justice, et le dispositif pourrait effectivement être amélioré. Cet amendement va plus loin qu'une simple suppression de l'obligation alimentaire. Outre la suppression de l'obligation d'aliment des enfants

à supprimer la possibilité pour le juge de maintenir une obligation d'aliment lorsqu'il prononce un retrait total d'autorité parentale. Or le retrait total d'autorité parentale couvre bien d'autres cas que les violences conjugales, tels que l'alcoolisme du parent ou le défaut de soins. Il n'y a donc pas de raison de supprimer cette souplesse, sachant de surcroît qu'en cas de meurtre ou de violence sur l'autre parent, le juge ne fera pas juge ne fera pas usage de cette possibilité. Par ailleurs, cet amendement tend à supprimer la possibilité pour le parent dont l'autorité parentale a été retirée d'en demander le rétablissement en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat sur l'autre parent. Une telle disposition inclurait toute possibilité pour un juge

: La parole est à M. Jean-Pierre Grand. Dans les restitutions du groupe de travail « justice » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de décharger les enfants de l'obligation alimentaire envers le parent condamné pour homicide volontaire sur l'autre parent. Le code civil prévoit que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. En cas d'atteinte volontaire à la vie par le conjoint, il est proposé de permettre aux juges

qui prévoit qu'en cas de meurtre ou assassinat d'un parent par l'autre, la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale du meurtrier. Il s'agit d'ajouter que la juridiction pénale se prononce également sur le maintien ou non de l'obligation alimentaire de l'enfant vis-à-vis du parent criminel survivant. Cet ajout semble inutile, car, en cas de meurtre, le retrait prononcé est total, ce qui entraîne automatiquement une dispense de l'obligation alimentaire en application de l'article

Josiane Costes. La dernière réforme du divorce a introduit le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, afin de désengorger les tribunaux pour les divorces non conflictuels. Celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'un des deux époux bénéficie d'une ordonnance de protection contre l'autre. Cet amendement vise donc à exclure explicitement cette possibilité dans la loi.

Mme Françoise Cartron. Cet amendement a pour objet de suspendre l'exercice de l'autorité parentale en cas d'homicide volontaire par le conjoint, sans qu'il soit besoin d'une décision du juge, et ce dès la phase d'enquête ou d'instruction. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l'intérêt de l'enfant le commande. Comme le Grenelle des violences conjugales nous y invite, cette rédaction vise ainsi à indexer notre droit sur le réel lorsqu'un père commet des violences sur la mère de ses enfants, la plupart du temps en face de ces derniers, on peut légitimement supposer que la relation qui les lie est fortement dégradée, au moins le temps du jugement de la procédure. Ainsi, maintenir envers et contre tout le lien physique entre un enfant et son père ne semble raisonnable ni pour l'enfant ni pour la mère, qui est mise en péril dès qu'elle exerce son droit

Cet amendement traduit une recommandation formulée par la délégation aux droits des femmes dans plusieurs de ses travaux sur les violences faites aux femmes. Il vise à favoriser un changement de regard sur la question de l'autorité parentale, afin de rendre plus évidente la suspension, voire le retrait

à l'occasion des droits de visite et d'hébergement des enfants. Il est donc urgent de favoriser la réflexion sur un aménagement facilité de l'autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, comme l'a d'ailleurs annoncé le Premier ministre dans le cadre du lancement du Grenelle des violences

la question de l'autorité parentale et de son maintien en cas de violence intrafamiliale est au coeur de nos débats. C'est une préoccupation vive, qui a fait l'objet d'annonces du Premier ministre et du Gouvernement depuis quelques mois. Le travail est en cours, et le rapport permettra au Parlement d'en être utilement tenu informé et de connaître quelles pistes sont explorées. La commission est donc favorable à cet

tenter de lui donner la mort, ou avoir volontairement porté des coups ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Cet amendement vise à exclure également de la succession le conjoint qui a été condamné à une peine criminelle pour avoir commis des violences envers le défunt, même si celles-ci n'ont pas entraîné sa mort. Les faits sont suffisamment graves pour entraîner une indignité successorale. L'automaticité permettrait de mettre fin à des situations choquantes. Par ailleurs, la victime conserverait toujours la possibilité de confirmer sa volonté de maintenir son conjoint dans sa succession, en application de l'article 728 du même code. Quel est l'avis du Gouvernement

à créer une exception légale aux droits de succession du conjoint qui est condamné à une peine criminelle pour des faits de violence. Aujourd'hui, les causes d'indignité successorale sont prévues lorsque l'auteur des faits est directement responsable du décès de la victime.

pour avoir commis des violences envers le défunt, même si cela n'a pas entraîné la mort de ce dernier. La décision d'exclure le conjoint de la succession serait prononcée par le tribunal. Par ailleurs, la victime conserverait la possibilité de confirmer, de son vivant, sa volonté de maintenir son conjoint dans sa succession, en application de l'article 728 du code civil.

L'article 5 prévoit, lors du dépôt de plainte, l'information de la victime de violences conjugales sur ses droits à bénéficier du dispositif de protection électronique. La commission des lois a adopté une rédaction de compromis prévoyant que cette information se ferait de manière orale et par la remise d'un document. la prise en charge et l'information sont primordiaux en la matière, les officiers et agents de police judiciaire qui reçoivent la plainte ne peuvent pas connaître tous les dispositifs spécifiques applicables à l'ensemble des crimes et délits. Cette difficulté est renforcée par l'ajout en commission de l'obligation d'information sur la possibilité de bénéficier de l'ordonnance de protection. Il est donc proposé de préciser que l'information de la victime s'effectuera par la remise d'un document l'informant de ses droits. Cette solution permettra d'offrir une réponse complète et uniforme sur l'ensemble du territoire. Bien évidemment, la victime venue porter plainte pourra toujours être réorientée vers un agent mieux formé et plus apte à répondre à l'ensemble de ses interrogations. Une telle mesure a été restitutions du groupe de travail « accueil en commissariat et gendarmerie » du Grenelle des violences conjugales, qui prévoient notamment de remettre systématiquement un document d'information simplifié aux victimes, de « protocoliser » l'accueil des victimes dans les services de police et unités de gendarmerie et de renforcer les formations initiales et continues des forces de l'ordre. est l'avis de la commission ? Cet amendement traite des modalités d'information de la victime. La commission est favorable à ce que la victime reparte avec un document lui permettant de retrouver toutes les informations qui lui ont été présentées, mais ne souhaite pas que l'information se résume à la remise de ce document, qu'elle ne lira peut-être pas ou ne comprendra peut-être pas. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité préserver une information

la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La victime de violences conjugales est très fréquemment réticente à déposer plainte contre son conjoint violent. Elle privilégie bien souvent la main courante ou le procès-verbal de renseignement judiciaire. Même si le retrait d'une plainte n'éteint pas les possibilités de l'action publique, il est proposé d'aggraver les peines encourues par un conjoint violent.

j'aurais souhaité que l'évolution de notre droit en matière d'inceste soit discutée de nouveau aujourd'hui, dans la continuité de mes propositions antérieures sur le sujet, notamment lors de l'examen du précédent projet de loi soutenu par Mme Schiappa. Les violences sexuelles sont en effet une forme particulière de violence qui sévit parfois malheureusement au sein des familles. L'ensemble de ces amendements vise notamment à renforcer la qualification pénale des actes incestueux sur mineurs en créant une infraction spécifique pour les viols et agressions sexuelles incestueux sur mineurs. Il s'agissait de s'assurer que l'existence d'un acte incestueux d'un majeur sur un mineur de la même famille suffit à caractériser à elle seule la violence et la contrainte mentionnée à l'article 222-22 du code pénal, la notion de consentement en matière d'inceste n'ayant absolument aucun sens. visent à ce que tous les actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, soient considérés comme des viols ou des agressions sexuelles. Le droit positif en matière d'inceste prend en compte les « ascendants et les personnes ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait Ces nouvelles dispositions permettraient de prendre en considération non seulement les ascendants, mais aussi toutes les personnes mentionnées à l'article 222-31-1 du code pénal relatif à la qualification incestueuse des viols et agressions sexuelles. De plus, il n'y aurait plus besoin de démontrer l'autorité de droit ou de fait, l'inceste sera qualifié et puni de façon automatique, par le constat de la filiation.

parole est à M. Jean-Pierre Grand. Adopté en séance à l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du Gouvernement, l'article 7 prévoyait d'améliorer le dispositif du logement d'urgence en demandant aux préfets d'identifier des logements de droit commun pour attribution en urgence aux femmes victimes de violences. Au-delà d'être dépourvu de toute portée normative, cet article semblait être doublement satisfait à la fois par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose déjà que les femmes victimes de violences font partie des publics prioritaires pour l'attribution d'un logement locatif social et par l'expérimentation prévue à l'article 7 de la présente proposition de loi permettant de mettre rapidement des logements à disposition pour les femmes victimes de violences. La commission des lois a donc procédé à sa suppression. En effet, la sensibilisation des préfets passe essentiellement par les circulaires comme celle du 8 mars 2017 relative à l'accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté. Néanmoins, afin de renforcer

Mme Annick Billon. Aujourd'hui, certaines victimes de violences conjugales sont dans l'incapacité de se soustraire à leur agresseur, et ce alors même qu'il a été condamné, ce dernier continuant de faire peser des menaces sur son conjoint ou ex-conjoint et sur ses enfants. Cet amendement vise donc à assouplir les modalités de changement d'identité, afin de prendre en compte la situation particulièrement éprouvante des victimes de violences conjugales dont le cas ne semble pas entrer dans les critères actuels de changement de nom

Je m'interroge également sur le champ visé par cet amendement : si l'objet mentionne les victimes de violences conjugales, le dispositif fait référence aux victimes sans autre précision, ce qui est beaucoup plus large. Actuellement, l'identité d'emprunt peut bénéficier à des personnes victimes d'un réseau de proxénétisme ou de traite des êtres humains ou à des repentis qui ont empêché la réalisation d'un crime ou d'un délit. Ces personnes peuvent craindre des représailles de la part de la part de criminels agissant en bande organisée. Il est vrai que certaines victimes de violences conjugales peuvent redouter d'être victimes de représailles de la part de leur conjoint, notamment au moment du dépôt de plainte. Il nous semble cependant que le bracelet anti-rapprochement leur offre une protection plus appropriée

Cet amendement est déjà satisfait par la possibilité pour tout patient de demander la non-divulgation de sa présence à l'hôpital. Cette demande peut être faite lors des formalités administratives à l'accueil ou dans le service d'hospitalisation lors de l'admission. L'obligation de discrétion professionnelle qui s'impose aux professionnels de santé doit suffire à protéger la personne qui ne veut pas que sa présence à l'hôpital soit connue. Demande de retrait ou avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis. Madame Billon,

M. Jean-Pierre Grand. Dans les restitutions du groupe de travail « violences psychologiques » du Grenelle des violences conjugales, il est proposé de créer une incrimination du suicide forcé comme circonstance aggravante. Le code pénal prévoit que le fait de provoquer le suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Il est proposé de porter ces peines à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la provocation a conduit au suicide de son conjoint ou ex-conjoint.

lié par un pacte civil de solidarité sur celle qui est prévue pour le suicide d'un mineur. Il s'agit de répondre aux cas de suicides forcés. Cependant ce n'est pas nécessairement par la provocation directe au suicide que la victime est poussée à l'acte, mais tout aussi bien par le harcèlement moral. Il n'est donc pas sûr que cet amendement atteigne l'objectif

comme le montre le, qui, depuis 2015, le définit comme « le meurtre d'une femme en raison de son sexe ». Pourquoi susciter une réflexion sur la prise en compte de cette notion dans le code pénal ? Le meurtre d'une femme par son compagnon est un crime spécifique pour diverses raisons. il relève d'une vision de la femme considérée comme la propriété de son compagnon, qui ne supporte pas qu'elle le quitte, voire l'idée même qu'elle puisse lui échapper. Ensuite, le meurtre d'un conjoint peut avoir des conséquences terribles sur plusieurs générations. terribles sur plusieurs générations. S'il peut être perpétré par une femme sur un homme, on sait qu'une telle circonstance est extrêmement rare et que les victimes de mort violente au sein des couples sont, dans leur immense majorité, des femmes.

de féminicide dans le code pénal. Nous sommes traditionnellement réservés face aux demandes de rapports, qui ne sont pas toujours remis ou dont le contenu est décevant. Nous considérons de plus que le Parlement a les moyens de se saisir d'un sujet qu'il souhaite approfondir, en confiant à l'une de ses commissions ou délégations le soin

par un homme ou par une femme. J'observe qu'aucune des personnes que j'ai entendues n'a fait état d'un vide juridique qui empêcherait de sanctionner avec toute la sévérité requise le meurtre ou l'assassinat d'une femme par son conjoint.

On le sait, notre code pénal réprime déjà de façon spécifique et aggravée les meurtres commis à l'encontre de femmes, que l'on pourrait donc sociologiquement qualifier de féminicides. C'est le cas des meurtres qui sont commis en raison du sexe de la victime, commis au sein du couple, commis après un viol, une agression sexuelle ou une mutilation sexuelle, ou commis en raison d'un refus de mariage forcé par la victime. Dans l'hypothèse d'une aggravation de de la répression, faut-il qualifier ces crimes de féminicides ? Une telle réforme serait évidemment sans portée juridique, dans la mesure où la qualification de féminicide n'emporterait pas une aggravation de la peine encourue puisque le meurtre commis par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un est déjà puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Je rappelle d'ailleurs que la notion de parricide a été supprimée lors de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, et que celle d'infanticide n'a jamais été consacrée par la loi pénale. Enfin, cela pourrait être perçu comme une discrimination portant atteinte au caractère universaliste de notre droit. Il faudrait par ailleurs être suffisamment précis dans la définition juridique du concept, afin d'éviter des difficultés similaires à celles qui ont présidé à la reconnaissance de l'inceste pour laquelle, vous le savez, le Parlement a dû légiférer à deux reprises, en 2010 puis en 2016, à la suite de l'annulation des dispositions

C'est effectivement un sujet très important. En effet, aujourd'hui le juge aux affaires familiales peut accorder l'admission provisoire de la victime à l'aide juridictionnelle. En pratique la victime n'en bénéficie qu'à compter de la délivrance de l'ordonnance de protection, alors qu'elle en aurait besoin dès le stade de la demande. demande. La saisine par assignation, qui est plus rapide, a un coût. Certaines victimes n'ont pas les moyens de le financer. Dans ces conditions, l'octroi de plein droit de l'aide juridictionnelle aux demandeurs d'une ordonnance de protection me semble une idée intéressante pour accélérer le délai de délivrance de l'ordonnance de protection.

Il y a plusieurs manières de les aider financièrement. Soit nous considérons que toute femme qui dépose une plainte ou va devant une juridiction pour obtenir réparation de son préjudice ou protection

Les Républicains, et Naïma Moutchou, du groupe LaREM -qui ont rendu un rapport sur ce sujet. J'ai promis que nous aboutirions à une solution sur cette question de l'aide juridictionnelle dans l'une ou l'autre des formes que je viens d'évoquer avant le

est à Mme le rapporteur. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du pays du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil et de droit commercial, la collectivité de Nouvelle-Calédonie est compétente en matière civile. Il n'est donc pas justifié de prévoir que les articles 1 à 2 , relatifs au droit civil, s'appliquent dans cette collectivité. Le présent amendement vise donc à modifier en conséquence l'article 12. Quel est l'avis du